La séance est reprise. Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour un nouveau pacte ferroviaire. Je rappelle que la discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte

J'espère me tromper, mais je ne peux m'empêcher de penser que ce gouvernement, ou la prochaine majorité, pourrait procéder à une privatisation en recourant à une augmentation du capital. Ce n'est pas possible ... Je me répète, mais l'argument de la dette qui devrait être reprise par l'État, sans qu'aucune modalité de reprise ne soit évoquée mis à part un « on va se débrouiller » peu rassurant, serait un alibi parfait pour détruire le service public ferroviaire et le privatiser. C'est d'ailleurs très exactement ce qui a été fait pour France Télécom : transformation en SA en 1996, ouverture du capital en 1997, privatisation partielle en 2004 et fin de la minorité de blocage de l'État en 2007. Une décennie, c'est tout ce qu'il a fallu pour passer d'un organe public à un organe privé, mettant fin à cent quinze ans de téléphonie publique. Et quand on voit les inégalités de couverture téléphonique entre les territoires et la qualité du service, l'argent public déboursé pour pallier les manquements du privé, il y a de quoi être nostalgique Madame la ministre, au regard du passif, vous comprendrez aisément que le blanc-seing que vous nous demandez est inacceptable à nos yeux. La parole est à M. Fabien Gay,

de dividendes à ses actionnaires. Que s'est-il passé pendant cette période ? Les dividendes ont explosé, les conditions des salariés ont été dégradées et le prix du gaz a augmenté de 40 % en dix ans. Ce n'est donc pas une crainte.

Magner, sur l'article. Madame la ministre, vous participez à un gouvernement qui a engagé une importante réforme du rail et vous voulez aller vite. Certes, les objectifs affichés pour cette réforme ferroviaire sont ambitieux. En même temps, il s'agit de repenser l'organisation actuelle de la SNCF, d'améliorer son efficacité industrielle, de réduire ses coûts et de préparer l'entreprise publique à l'ouverture à la concurrence. ce nouveau pacte ferroviaire est issu des recommandations contenues dans le rapport que M. Spinetta a remis au Premier ministre le 15 février dernier. Élu du Puy-de-Dôme, je ne puis qu'exprimer mon inquiétude sur l'une des conclusions du rapport de M. Spinetta, celle qui concerne le déficit des lignes moins fréquentées. La tendance est claire : les lignes à grande vitesse vont continuer à être privilégiées au détriment des lignes qui constituent pourtant des éléments essentiels de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, l'Auvergne est toujours la seule région de France à n'être pas reliée à Paris par un train à grande vitesse. Longtemps, il a été promis la création d'une ligne à grande vitesse qui relierait Clermont-Ferrand à Paris en passant par Orléans et à destination de Lyon. Dans cette attente, les travaux pourtant nécessaires pour l'amélioration de la ligne Intercités ont été différés, les tronçons de ligne à plus de 200 kilomètres par heure prévus dans les contrats de plan successifs n'ont jamais été réalisés, si bien qu'il faut encore plus de trois heures- parfois trois heures vingt -pour parcourir les 400 kilomètres qui séparent Clermont-Ferrand de Paris.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, même si elle accepte le principe de l'ouverture à la concurrence dont j'aurai l'occasion de parler à d'autres moments,

? Nullement, puisque, à partir du moment où ces structures sont des SA, fussent-elles de capitaux publics, elles sont liées à l'accès au marché dans des conditions où l'État n'est plus garant de leur dette et, par conséquent, elles empruntent plus cher.

et on nous expliquera ensuite que, pour investir, il faut aller chercher de l'argent ailleurs. Où ? Dans le secteur privé. Ainsi, la boucle est bouclée. Boucle négative : nous avons besoin d'un service public fondé sur une entreprise totalement publique, car aucun profit dans les transports ferroviaires ne doit aller ailleurs qu'au transport ferroviaire péréquation tarifaire, aménagement du territoire, avenir de la SNCF.

Nous sommes opposés à ces changements de statut qui ouvrent la voie à la privatisation de la SNCF, et ce malgré toutes les subtilités d'écriture, quand bien même on indique que le capital est détenu intégralement par l'État et, par un ajout en commission, qu'il est incessible. En effet, si ces précautions sont bienvenues, elles ne changent rien sur le fond. L'ouverture du capital sera de toute manière toujours possible par le recours à une augmentation du capital et l'émission de nouveaux titres. La privatisation sera, de fait, facilitée par ce changement de statut, puisqu'une simple loi pourra revenir sur ces engagements de maîtrise à 100 %.

EDF, GDF, France Télécom ... Les managements ont évolué, pour se tourner vers les techniques du privé : rentabilité, clients, retour sur investissement ... tout un vocabulaire qui a accompagné la dégradation des services publics. Nous ne voulons pas d'un dessein identique pour l'opérateur ferroviaire. En quoi la forme serait-elle un obstacle à l'exercice des missions de l'opérateur public ? C'est tout l'inverse : elle permet aujourd'hui l'existence de prérogatives de puissance publique, par exemple l'insaisissabilité des biens ou encore, par la garantie de l'État, le recours à des taux intéressants, parfois même négatifs. La réforme menée en 2014 a conduit à préconiser un cadre, compatible avec les injonctions européennes, dans lequel la forme publique des entreprises pouvait être préservée. Pourquoi y revenir aujourd'hui ?

Nous pensons au contraire qu'il convient, au regard de la nature même des missions d'intérêt général qui incombent au système ferroviaire, de travailler aux complémentarités et à une intégration plus grande garantissant totalement et de manière pérenne le caractère public de l'opérateur au travers d'un statut spécifique. Pour cette raison, nous vous proposerons des amendements visant à supprimer ce passage en société anonyme, délétère et dangereux pour l'avenir du service public ferroviaire dans l'ensemble de notre pays. La parole est à M. Ronan Dantec,

À partir de 1989, les choses ont commencé à changer doucement. Certes, nous avions changé de majorité, la gauche avait repris la ville, mais, surtout, 1989, c'est l'arrivée du TGV à Nantes et cela correspond à la création progressive de cette métropole, qui est aujourd'hui l'une des plus attractives de France et d'Europe. Le TGV a profondément modifié le territoire français. Il a permis un début de rééquilibrage par rapport à ce que l'on appelait « Paris et le désert français ». La société française

de la métropole comme seul moyen de rééquilibrage du territoire, même si on voit encore avec l'arrivée du TGV à Bordeaux à quel point cela modifie le territoire. Ce qui se joue maintenant, ce sont les territoires autres. Dans ces territoires autres, le train jouera probablement le même rôle de rééquilibrage. Par conséquent, il faut non pas se priver de la capacité d'aménagement du territoire

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la répétition est l'un des piliers de la pédagogie. L'article 1 A prévoit le passage en société anonyme à capitaux publics de SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau.

L'argument consistant à expliquer que l'État doit se protéger de lui-même en limitant sa capacité à imposer des choix politiques coûteux à la SNCF a peu de portée. Celui qui prône une plus forte intégration du groupe ne vaut pas davantage.

un outil au service éventuel d'une libéralisation du service public ferroviaire français, bien au-delà des exigences européennes. La création par la loi de 2014 d'un groupe ferroviaire unifié composé de trois EPIC traduisait un compromis à la fois juridique et social, en accord avec avec les règles européennes. Oui, le statut de SA est la forme juridique la mieux adaptée pour une entrée en bourse. Il ouvre la possibilité d'une privatisation. GDF ou France Télécom en sont des illustrations. Comment ne pas imaginer demain

un passage d'EPIC en SA entraînera une dégradation de la part des agences de notation. La société anonyme est solidaire de ses dépenses excessives, à concurrence des capitaux propres de la société. Sans garantie de l'État, la nouvelle société n'aura pas les mêmes capacités d'endettement, les emprunts seront plus difficiles à lever La transformation en 2004 d'EDF en SA n'a pas empêché la dette de la nouvelle SA de déraper. À tout le moins et pour conclure, madame la ministre, quel intérêt à transformer en société anonyme SNCF Réseau, qui, par nature, ne peut qu'être en situation de monopole ? L'exemple du Royaume-Uni, qui a renationalisé

est à Mme la ministre. J'entends que l'on puisse vouloir parler d'une autre réforme que celle que l'on est en train de mener. Néanmoins, il faudra prendre le temps de parler aussi de la réforme que le Gouvernement a proposée. Une autre réforme de privatisation et de démantèlement, une autre réforme de désengagement de l'État ? Ce n'est pas cette réforme qui est proposée par le Gouvernement ! Vous posez la question de la transformation des EPIC en SA.

conduit à une avancée pour le transport ferroviaire depuis 1982 ? Regardez les chiffres ! Regardez les courbes ! C'est précisément à partir de ce moment-là que la dette de la SNCF a commencé à augmenter. Si la SNCF avait eu un autre statut, personne n'aurait pu se permettre d'en laisser filer ainsi la dette. C'est à partir de ce moment-là, aussi,

de la succession de réformes imposées au rail français au cours des dernières années, sous couvert de le rendre plus performant : privatisation du fret ; mise en concurrence du trafic de voyageurs ; découpe de la SNCF en une myriade de filiales de droit privé, qui, souvent, se concurrencent ; recours à des personnels sous-payés, subissant les mêmes entorses au droit du travail que les salariés de Veolia Cargo ou d'Euro Cargo Rail, filiale de la madame la ministre, le scénario est assez clair, et la rédaction de cet article 1 A ne manque pas de sel. Ainsi, outre le passage au statut de SA, vous renforcez sous couvert d'unification la filialisation du groupe SNCF, filialisation qui transformera la SNCF en coquille vide tous les actifs seront transférés vers les filiales. Dès lors, la règle de l'incessibilité de son capital n'est qu'un leurre toujours à l'article 1 A, que la création de filiales par la SNCF ne portera pas atteinte à l'application du statut, ainsi que des accords et conventions collectives. Pourtant, la SNCF compte plus de 1 000 filiales, lui ayant permis de supprimer plus de 30 000 emplois sous statut depuis 2002. Plus d'un quart de ces suppressions d'emplois ont concerné la gestion de la maintenance des infrastructures ferroviaires, soit l'équivalent de 30 usines Molex

traitons du domaine public ferroviaire et il existe un principe de niveau constitutionnel selon lequel le domaine public appartient à une personne publique. Voilà encore un procès inutile : le domaine public appartient à une personne publique ; ça tombe bien, puisque la SNCF est une société publique

monsieur le président

ni caricature, ni chiffon rouge ! Je voudrais attirer l'attention de la représentation nationale sur le fait que nous sommes attendus, je l'ai dit il y a quelques instants dans la discussion générale. Nous sommes attendus et nous sommes regardés.

soit vous êtes en train de nous expliquer que le choix de la société anonyme vous donne des libertés pour l'avenir, et c'est bien ce qui nous fait peur ! La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

faire sauter le verrou du statut d'établissement public pour pouvoir privatiser dans un second temps. Souffrez que nous ne soyons pas d'accord.

Madame la ministre, vous dites qu'un des avantages du statut proposé serait de conférer plus d'unité à l'ensemble de l'entreprise ferroviaire ainsi constitué. Je partage cet argument.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

Si le projet de loi prévoit que le capital social de la SNCF sera détenu intégralement par l'État et incessible, nous avons de bonnes raisons de penser que l'abandon du statut d'EPIC ne constituera qu'une première étape vers une ouverture ultérieure du capital des nouvelles SA. Souvenons-nous, mes chers collègues, de ce qui s'est passé dans d'autres secteurs économiques, comme ceux des télécommunications ou, cela a été rappelé, de l'énergie. Nous estimons donc que le statut d'EPIC constitue le meilleur rempart contre une privatisation éventuelle. Il nous prémunit ainsi contre toute ouverture de capital. Il interdit le versement de dividendes aux actionnaires, en l'occurrence, à l'État. Il offre la garantie illimitée de pouvoir recourir à des emprunts à des taux d'intérêt bas, bien inférieurs à ceux qui sont pratiqués sur les marchés financiers. L'enjeu, madame la ministre, est de pérenniser la maîtrise publique du service public des transports, de maintenir Gares & Connexions dans le giron de SNCF Réseau et d'empêcher la filialisation, à terme, de cette activité.

en société nationale ne conduira pas à la privatisation de la SNCF ne nous convient pas. D'autant qu'il ne s'agit pas là d'une innovation et que nous avons la preuve, par l'histoire, que cela ne se fera pas dans le sens de l'amélioration du service des usagers ni de la santé économique de l'entreprise. En effet, comme nous l'avons indiqué dans l'objet de notre amendement, le mouvement de transformation des EPIC nationaux en sociétés anonymes

Plus révélateur encore de la pente abrupte vers la privatisation et de la casse sociale annoncée, on peut citer l'exemple de l'ancienne entreprise publique SEITA, fondée en 1926, devenue EPIC en 1959, puis société nationale en 1980, avant d'être privatisée en 1995, entraînant une série de fermetures d'usines avant son rachat par Imperial Tobacco, dont elle est devenue filiale avec, à la clé, un plan social de grande ampleur et la suppression de 2 440 emplois en Europe. Je ne reviendrai pas sur les autres transformations en société anonyme que nous avons déjà évoquées : TDF, La Poste, France Télécom, ou encore GDF, EDF et, bientôt, Aéroports de Paris. L'argument expliquant cette évolution est bien connu, à force d'avoir été répété ces établissements paraissent de nos jours atteints d'une malformation congénitale, leur caractère trop public, qui les rendrait inadaptés au secteur d'activité dans lequel ils évoluent, soit parce qu'ils sont gênés par les pesanteurs administratives, soit parce qu'ils tirent de leur attachement à l'État des avantages économiques à l'égard de leurs concurrents. Permettez-nous de vous rappeler la définition d'un EPIC, afin de préciser de nouveau en quoi il est absolument nécessaire de conserver ce régime juridique pour ce secteur d'activité essentiel qu'est le ferroviaire que ce soient des créations pures ou des nationalisations anciennes, comme c'est le cas pour la SNCF, la personne morale de droit public que représente l'EPIC a pour but la gestion d'une activité de service public, dont le bon fonctionnement est essentiel compte tenu de la spécificité du service public à assurer, une entreprise industrielle ou commerciale privée soumise à la concurrence ne peut pas être aux manettes. C'est la raison même de l'existence des EPIC.

comme son caractère public, est le garant d'un maillage territorial efficace et remplit aujourd'hui un rôle tout aussi social qu'économique, lui permettant de concourir à la solidarité nationale. Avec la libéralisation et le changement de statut, c'est la nature même du service public qui est mise en cause. social, car le rail est un rappel de l'État dans des zones qu'il a parfois abandonnées. Quand vous habitez dans un territoire enclavé, le train constitue souvent le dernier service public accessible et le moyen de se rapprocher des zones les plus denses. En cela, le réseau ferré est un outil structurant du territoire de la République. social, aussi, car le rail constitue, pour de nombreuses personnes, le seul moyen de locomotion possible. L'avion est beaucoup plus cher et d'un accès plus éloigné, et la voiture demande des investissements importants. Il ne reste alors plus que le train. économique, enfin, car les entreprises ont tout intérêt à avoir un réseau ferré efficace, faisant l'objet d'un investissement public massif, pour transporter facilement et de manière performante leurs salariés et leurs marchandises. Outre ces éléments, on ne peut omettre les enjeux environnementaux du réseau ferré. Le Grenelle de l'environnement verra-t-il ses objectifs suivis par la France en matière de part modale du non-routier et du non-aérien ? Alors que, d'après un rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, de l'exposition à l'ozone et aux particules, il est urgent de revaloriser le moyen de transport le moins polluant dans notre pays. De par son rôle structurant et son caractère universel, le rail doit faire l'objet d'un fort investissement public, mais il est nécessaire de rappeler qu'il est l'affaire de toutes et de tous, et un acteur majeur de la solidarité nationale. Quand nous entendons des éditorialistes avancer, sans aucun recul, que « la SNCF coûte 1 000 euros à chaque Français, même ceux qui ne prennent pas le train je me demande si leur position est la même en ce qui concerne l'éducation nationale, la sécurité sociale, les aides à la presse, pour celles et ceux qui ne scolarisent pas leurs enfants, ne sont pas malades et ne lisent pas

La part modale du ferroviaire dans le transport de marchandises est en effet passée de 10,6 % en 2015 à 9,6 % en 2017. Au regard de ces chiffres inquiétants, le développement du transport ferroviaire demeure un enjeu considérable et nécessite qu'une stratégie de promotion des modes de transport verts soit inscrite dans le droit. Le verdissement de nos modes Le verdissement de nos modes de transport est un objectif de court terme, essentiel à nos politiques de développement durable et de préservation de l'environnement. C'est un sujet sur lequel nous nous battons tous depuis un certain nombre de mois.

comment comptez-vous mettre la SNCF et son développement au service de la transition écologique, dont notre pays a absolument besoin pour respecter les accords conclus dans le cadre de

En effet, depuis plusieurs années, nous assistons à une externalisation des activités stratégiques en dehors de l'EPIC. On dénombre ainsi, non pas 900 filiales, monsieur Émorine, mais plus de 1 000

concurrencent aujourd'hui directement des branches ou secteurs d'activité de l'EPIC. Si nous comprenons la volonté de croissance de la SNCF, voire d'une diversification de ses activités, cette dernière ne peut s'entendre que par la volonté de renforcer l'offre aux usagers, et non de mettre en place une concurrence intragroupe. Ainsi, à l'heure actuelle, si des filiales peuvent venir concurrencer l'activité principale de la SNCF, de SNCF Réseau ou de SNCF Mobilités, cela ne semble pas cohérent, y compris au regard de l'importance des missions de service public remplies par la SNCF en termes d'aménagement du territoire ou de transition écologique. Nous demandons donc, non pas d'interdire la possibilité pour la SNCF, SNCF Réseau ou SNCF Mobilités de créer des filiales, mais simplement d'en limiter le champ aux activités qui ne sont pas du ressort des trois sociétés constituant le groupe ferroviaire, afin d'éviter une concurrenceintragroupe. Nous proposons également, dans le même sens, de restreindre la faculté de création de filiales aux activités non ferroviaires ayant un objet connexe et complémentaire aux missions de l'ensemble

filiales. On peut imaginer la création de filiales régionales si une autorité organisatrice l'exige dans le cadre d'attributions directes ou de mises en concurrence. Dès lors, pour assurer la cohérence sociale du groupe public ferroviaire, en particulier une politique de gestion des ressources humaines dynamique, offrant des possibilités de parcours professionnels attractifs, il apparaît essentiel d'anticiper ces possibles évolutions, et de prévoir que les filiales ferroviaires ainsi créées restent dans le périmètre du groupe public ferroviaire.

de l'énergie ou des télécommunications, le même processus de transformation s'est traduit par l'ouverture du capital des EPIC transformés en SA, à l'exemple de la filiale gestionnaire des infrastructures de transport d'électricité à haute tension, RTE.

Christine Prunaud. Par cet amendement, nous nous opposons à la filialisation de Gares & Connexions, qui est aujourd'hui une direction intégrée à l'EPIC SNCF Mobilités. La question de la filialisation ou de la privatisation des gares n'est pas nouvelle. Gares & Connexions, c'est la gestion et la rénovation d'un patrimoine de près de 3 000 gares sur le territoire national, la gestion de revenus immobiliers, le premier accès à la ville, la garantie d'une desserte fine de notre territoire. Gares & Connexions représente aussi des enjeux de mobilité, de fluidité, de sécurité. Ce n'est pas une vue de l'esprit : le démantèlement des gares de proximité constitue l'un des effets concrets de la privatisation du secteur ferroviaire menée à l'échelle européenne depuis un quart de siècle. D'autres choix que la filialisation sont possibles. Ainsi, le rapport précise qu'il serait envisageable de rattacher Gares & Connexions à SNCF Réseau sous forme de direction dédiée, « aurait l'avantage de simplifier la gestion patrimoniale des gares en réunissant l'exploitation des bâtiments des gares et celle des quais, et de créer un guichet unique pour l'accès des entreprises ferroviaires aux gares ». Ce serait un

qu'idéologique. Le choix de la filialisation, c'est le démantèlement du patrimoine ferroviaire, commun à tous nos concitoyens.

en société anonyme à capitaux publics, indépendante du groupe public ferroviaire, nécessiterait que lui soient affectés les bâtiments des gares et certains actifs de SNCF Réseau. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cette disposition.

une meilleure coordination au sein des gares et à ne plus s'interroger pour savoir si un réseau électrique appartient à l'une ou l'autre

Votre commission a voté en faveur d'une autonomie organisationnelle, décisionnelle et financière. Le Gouvernement partage cet objectif, à

de loi prévoit désormais que Gares & Connexions sera rattachée à SNCF Réseau sous la forme d'une filiale disposant d'une autonomie organisationnelle, décisionnelle et financière. Nous sommes opposés à cette filialisation et nous avons déposé des amendements en ce sens, qui n'ont malheureusement pas été adoptés. En effet, en droit des sociétés, une filiale est définie comme une société dont le capital est détenu à plus de 50 % par la société mère. Il y a donc,, constitution d'un capital. MM. Maurey et Nègre, auteurs de la proposition de loi sur la transposition du quatrième paquet ferroviaire que nous avons examinée voilà quelques semaines, prévoyaient que le capital de Gares & Connexions serait composé majoritairement de capitaux publics. Nous souhaitons, par précaution, que le capital de cette nouvelle filiale soit détenu intégralement par des capitaux publics de l'État, et- pourquoi pas ?-des collectivités territoriales, parties prenantes à l'avenir des gares. L'amendement n° 237,

organisationnelle, décisionnelle et financière. Le rapporteur a également conforté l'autonomie décisionnelle de Gares & Connexions en prévoyant un contrat entre la nouvelle filiale et l'État d'une durée de cinq ans, lequel portera en particulier sur divers objectifs de qualité de service, de trajectoire financière et d'investissement dans les gares. Vous avez aussi souhaité, monsieur Cornu, renforcer l'association des collectivités territoriales à la gouvernance des gares. C'est une bonne chose, et nous nous en félicitons. Nous souhaitons toutefois que, au sein du conseil d'administration de la filiale Gares & Connexions, figurent toutes les parties prenantes, qui pourront dès lors peser sur les orientations et décisions relatives à la gestion des gares. Cela nous semble indispensable si l'on filialise cette activité. L'amendement n° 129, présenté par M. Longeot,

dernières sont les portes d'entrée des villes et sont des lieux de vie. Quand on rénove une gare, c'est un quartier de ville qui se reconstruit. Des études ont montré que les investissements dans les gares créeraient des investissements supplémentaires grâce au travail partenarial avec les villes, les intercommunalités, les métropoles et les régions. En moyenne, un euro investi dans une gare entraîne quatre euros d'investissement dans le quartier de celle-ci. Il y a donc un effet de multiplicateur économique. Aujourd'hui, Gares & Connexions a prévu d'investir 1,5 milliard d'euros d'ici à 2020. Il faut non pas casser cette dynamique, mais au contraire l'accélérer. Il est nécessaire, dans le cadre de la réforme, de donner les moyens à la nouvelle filiale SNCF Réseau d'avoir les capacités d'investir davantage dans les gares et territoires. Gares & Connexions est une petite structure agile, peu endettée, dont l'activité est bénéficiaire. L'objet de cet amendement technique est de préciser que les comptes de SNCF Gares & Connexions seront mis en équivalence et non consolidés dans les comptes de SNCF Réseau. Cela signifie que les dettes de SNCF Réseau et de Gares & Connexions ne seront pas mélangées. En effet, la consolidation des comptes empêcherait Gares & Connexions de poursuivre la dynamique d'investissements dans les gares, car sa dette serait agrégée avec celle de SNCF Réseau, restera importante malgré le désendettement partiel. Réciproquement, les emprunts nécessaires au financement des gares alourdiraient inutilement la dette de SNCF Réseau.

Jacquin. Dans le même sens, au vu des nouvelles potentialités des gares dans les grandes villes- ces espaces devront conjuguer le ferroviaire, l'intermodalité et peut-être d'autres fonctions de service ou de commerce -, il nous semble intéressant d'élargir le conseil d'administration de ces gares. Nous proposons donc que les collectivités territoriales- villes, agglomérations, métropoles, régions -, mais aussi les usagers et les organisations syndicales puissent avoir un droit de regard sur les décisions relatives à la gestion

commerce. Ces espaces couvrent aujourd'hui 180 000 mètres carrés accessibles dans les gares et reliés au réseau de transports multimodaux. Nous proposons que des superficies puissent être réservées aux collectivités locales souhaitant les louer, afin de favoriser le développement d'activités à but non lucratif maisons de service public, activités associatives reconnues d'utilité publique, crèches, salles de réunion, etc. Les gares sont génératrices de flux de mobilité importants et sont des lieux névralgiques de passage régulier de nos concitoyens. Il est donc pertinent de réserver une partie de ces espaces publics aux collectivités territoriales. Cette zone est définie au cas par cas entre Gares & Connexions et les collectivités territoriales concernées. Il s'agit de réenchanter nos gares et de saisir l'opportunité de locaux au coeur des intermodalités qui puissent bénéficier à tous. Les gares sont notre patrimoine commun, héritage d'un investissement public

directe entre le gestionnaire de gares et l'État relative à la gestion des gares de voyageurs. Elle a aussi conforté l'association des collectivités territoriales à la gouvernance des gares de voyageurs. Pour autant, si les auteurs de l'amendement se félicitent de ces avancées, ils souhaitent également que les collectivités territoriales soient associées à tout projet concernant l'avenir des gares. L'amendement n° 36, présenté par Mme M. Guillaume Gontard. L'ambition de Gares & Connexions, y compris du fait de sa filiale, doit faire l'objet d'une vigilance de la puissance publique. À l'heure actuelle, seule l'ARAFER est saisie pour avis sur les projets de contrat et d'actualisation.

En effet, selon l'un des axes forts présentés par le Gouvernement ces dernières semaines, cette réforme est censée sécuriser une entreprise publique centrale et stratégique. Elle est centrale, car elle fait partie du quotidien de toutes et tous. Elle est stratégique, car ses implications dans la définition de toutes les politiques sont fortes. C'est tout le sens de cet amendement, qui vise à raffermir le contrôle de la représentation nationale sur un fleuron de notre pays. Il est d'autant plus dommageable d'avoir exclu le CESE du processus que sa nature même nous offre un regard expert sur toutes les questions liées au développement des gares. Je pense aussi à la question environnementale, ou encore, les gares pouvant faire office de commerces ou services à proximité des habitations, à la politique d'aménagement du territoire. Enfin, l'objet même des projets de contrat et d'actualisation nous oblige à la plus grande vigilance démocratique et à un contrôle efficace du Parlement. Il est regrettable de dénier à la représentation nationale toute intervention dans des projets de contrat définissant le paysage de nos villes et la qualité du service public national ferroviaire. L'amendement n° 74, présenté par Mme

nous craignons l'externalisation par la filialisation d'un certain nombre d'activités au sein de SNCF Mobilités, que ce soit le fret ou les trains express régionaux. Ce découpage de l'entreprise publique est contraire à l'idée même d'une meilleure cohérence dans le groupe ferroviaire et à une meilleure intégration. Ainsi, vous avez annoncé, madame la ministre, alors que la réforme était en cours d'examen à l'Assemblée nationale, la volonté du Gouvernement d'aller vers la filialisation du fret. Nous considérons que cette filialisation, qui a été repoussée par tous les gouvernements depuis plus de dix ans, est de très mauvais augure pour cette activité d'intérêt général. Vous soutenez aujourd'hui qu'elle permettrait une recapitalisation ; nous pensons au contraire que cette recapitalisation, certes utile et nécessaire, est possible sans faire de cette branche une société anonyme. En effet, en filialisant cette activité, vous la condamnez sur le long terme à l'équilibre, ce qui n'est ni possible ni souhaitable, quel que soit le montant des péages. Alors que le transport de marchandises par train ne représente que moins de 10 % du transport de marchandises global, nous estimons que la SNCF doit mener une politique, non pas de limitation de l'activité sur les axes les plus soutenables, mais au contraire de massification et de développement de l'offre, en relançant les triages. Comment est-il possible,

du fret signerait l'arrêt de mort de son développement. Soyons clairs, cette volonté de filialisation, que nous apprenons parfois par la presse lorsque celle-ci se procure des documents confidentiels, est le signe de la volonté du Gouvernement de s'engager dans la voie d'une privatisation

Nous prônons, pour notre part, une entreprise intégrée sous le modèle d'un EPIC, car c'est la forme juridique la plus aboutie pour l'exercice de cette mission de service public. Nous demandons donc, par cet amendement, la suppression de la possibilité de créer des filiales au sein de SNCF Mobilités.

parce que ce dernier ouvre la possibilité, pour le Gouvernement, de statuer sur les modalités de mise en place de conventions collectives différentes au sein de filiales, si la négociation collective n'a pas abouti dans un délai de six mois.

les niveaux de négociation collective adaptés aux différentes activités du groupe, cet amendement tend à conforter le principe de l'unité sociale qui consiste à garantir au sein de l'ensemble du groupe un même socle de droits. Afin de permettre notamment la mobilité professionnelle au sein du groupe et de préserver une forme de solidarité sociale, il est important de rappeler que ce socle doit avoir une large assise sans interdire la subsidiarité nécessaire.

est à M. Fabien Gay. Par cet amendement, nous souhaitons donner de la valeur à l'engagement du Gouvernement de faire des parts des sociétés anonymes créées par le présent projet de loi, en lieu et place des EPIC, des actions réellement incessibles.

qui s'est passé pour les autres fleurons industriels de notre pays qui ont été progressivement ouverts à la concurrence. Ce schéma est connu, il est simple. D'abord, la loi entérine le changement de statut, arguant de la souplesse et de la conformité au droit européen de la forme de société anonyme. À ce moment-là, le gouvernement en place promet, la main sur le coeur, que l'entreprise restera à 100 % publique.

Nous n'avons donc aucune foi dans vos promesses comme dans vos déclarations. Trente ans de libéralisme aveugle nous prémunissent- un peu ... -contre toute naïveté.

-d'une clause d'inaliénabilité, afin de rendre les actions véritablement incessibles. Vous le savez, toute société anonyme peut prévoir une telle clause pour une durée déterminée. Évidemment, cela ne nous prémunit pas contre les risques d'ouverture du capital par son augmentation, mais c'est une assurance qui serait bienvenue pour rassurer les organisations syndicales. La clause d'inaliénabilité a pour objet d'interdire la cession ou la transmission des droits sociaux sur lesquels elle porte. Elle permet le maintien des associés ou de certains d'entre eux pour assurer la pérennité de la société. Dans une société anonyme, une telle clause ne peut être justifiée que si elle repose sur un intérêt légitime. Nous considérons que, dans le domaine ferroviaire, le maintien d'un opérateur exclusivement public- étatique, plus exactement -constitue un intérêt légitime pour des raisons tenant à l'intérêt général que constitue le droit à la mobilité pour nos concitoyens.

Certes, il est indiqué dans le projet de loi que le capital des futures sociétés anonymes sera exclusivement détenu par l'État, mais nous estimons que cette disposition n'est pas suffisante pour garantir dans le temps la pérennité de cette maîtrise publique. Nous considérons nécessaire de verrouiller les statuts par des clauses spécifiques. Ainsi, après avoir proposé une clause d'inaliénabilité, nous proposons, par cet amendement, l'insertion dans les statuts d'une clause d'agrément. La clause d'agrément sert traditionnellement à contrôler et à stabiliser l'actionnariat d'une société. Elle permet de contrôler l'entrée de tiers au capital et, lorsque les cessions de titres entre associés ou actionnaires déjà présents sont concernées, de contrôler aussi la répartition des titres.

dans des proportions telles que les représentants de l'État ne disposent pas seuls de la majorité des voix. L'existence d'une telle clause permettrait une réelle consultation

et remet en cause les dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles régissant les situations des personnels employés par le groupe SNCF après la date du 1 janvier 2020. Or les personnels recrutés après cette date ne devraient pas être considérés comme des employés de seconde zone et le statut particulier des cheminots doit perdurer- n'en déplaise au Gouvernement et à ses considérations d'ordre idéologique

C'est donc uniquement la pression sur les salaires qui permettra une différenciation. C'est pourquoi les futurs employés ne seront pas fonctionnaires, ce qui passe par la destruction du statut des cheminots, afin que les personnes recrutées après 2020 relèvent du droit commun, celui qu'a créé la loi Pénicaud qui instaure un code du travail entreprise par entreprise ... En outre, vous ne parviendrez jamais à prouver que c'est le statut des cheminots ou le manque de concurrence qui est responsable des problèmes techniques

emprunts contractés sur les marchés financiers, ou encore, nous l'avons déjà dit, du désinvestissement de l'État. Pour conclure, une seule voie est envisageable et il est encore temps de faire machine arrière pour maintenir et améliorer le statut des cheminots dans le cadre d'une SNCF intégrée et publique.

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi indique que SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités remplissent des missions de service public. Cette formulation met déjà en lumière le rôle particulier de ces sociétés,

visent à préciser que le groupe public ferroviaire exerce ses missions dans le domaine du transport ferroviaire et de la mobilité, en poursuivant un objectif

Ces différentes propositions de rédaction montrent bien que l'on peut compléter à l'envi les objectifs assignés au groupe. Or les différents ajouts proposés peuvent être regroupés, à mon sens, au sein de l'objectif de

L'amendement n° 24 vise à préciser que les sociétés SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ne peuvent pas exercer d'activités qu'elles assurent déjà elles-mêmes par l'intermédiaire de filiales. Ce faisant, l'adoption de cet amendement interdirait, par exemple, à SNCF Mobilités d'exercer des activités de transport ferroviaire par le biais d'une de ses filiales comme Keolis. Ces filiales participent pourtant pleinement à la croissance des activités du groupe public unifié. L'avis de Dans la lignée du précédent, l'amendement n° 25 tend à ce que les filiales du groupe public unifié ne puissent exercer que des missions connexes et complémentaires à celles qui sont exercées par le groupe. Avis défavorable. 215 a pour objet d'élargir le périmètre du groupe public unifié, afin qu'il regroupe SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités, ainsi que l'ensemble des filiales de ces entités qui exercent une activité de de transport ferroviaire ou de marchandises ou une activité liée aux gares de voyageurs. Actuellement, le groupe public ferroviaire regroupe SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités. Cela a un sens, puisque ces trois entités forment une unité sociale elles emploient des salariés régis par le statut, dont les conditions de recrutement, de formation et d'évaluation professionnelles sont communes, et qui ont des instances représentatives du personnel qui mutualisées. Le projet de loi conserve cette unité sur le même périmètre

agissent dans des domaines variés, par exemple dans les secteurs du transport par autocar, de la logistique, de la gestion de parkings ... Bloquer toute possibilité d'évolution du capital de ces filiales est disproportionné et sans lien avec l'objectif poursuivi de maintenir le caractère public du groupe unifié. C'est pourquoi

dérogatoire. La rédaction de l'amendement va, en fait, à l'opposé de l'intention de ses auteurs, puisqu'elle fait du statut la dérogation à la règle que constituerait l'emploi sous le régime de la convention collective

n° 236 vise à préciser que le capital de Gares & Connexions sera détenu en intégralité par des capitaux publics. Sur la forme, cette rédaction est assez étrange : il conviendrait en effet d'indiquer que le capital est intégralement intégralement détenu par des personnes morales de droit public, et non par des capitaux publics- expression qui ne veut pas dire grand-chose. Sur le fond, autant je suis tout à fait d'accord pour prévoir que le capital de SNCF, de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau sera intégralement public et- cela a déjà été répété ... - incessible, autant cela se justifie moins pour le gestionnaire de gares qui exerce des activités de service public, comme l'accueil et l'information en gare, mais également des activités commerciales ou urbanistiques. Afin d'encourager le développement de ces activités et de favoriser les investissements en gare, il pourrait être utile que d'autres investisseurs puissent entrer au capital de Gares & Connexions, tout en garantissant que cette entité reste une filiale détenue en majorité par SNCF Réseau. L'avis est donc défavorable. L'amendement n° 237 tend à préciser la composition du conseil d'administration de Gares & Connexions, afin d'y prévoir la représentation des collectivités territoriales, des organisations syndicales et des associations d'usagers des transports.

cette méthode comptable doit permettre de faire en sorte que les emprunts nécessaires au développement des gares ne s'ajoutent pas à la dette de SNCF Réseau. Compte tenu de la difficulté à expertiser les conséquences de l'application d'une telle méthode, je m'en remets à l'avis du Gouvernement. du Gouvernement. L'amendement n° 238 vise la représentation des collectivités territoriales, des organisations syndicales représentatives et des associations d'usagers au sein des conseils d'administration des sociétés créées par Gares & Connexions pour gérer les espaces commerciaux des grandes gares. S'il me paraît nécessaire, bien sûr, d'associer les collectivités territoriales à la gestion des grandes gares sous ses différents aspects- investissements dans et autour de la gare, coordination des offres de transport, qualité de service ... il me semble en revanche disproportionné de prévoir leur représentation au sein des conseils d'administration de toutes les sociétés de gestion des espaces commerciaux en gare. Je vous propose d'en rester à rédaction de l'article 1 A, telle que modifiée par la commission qui, à travers la création de comités de concertation, a entendu renforcer l'association des collectivités concernées au pilotage des activités des grandes gares. L'avis est donc défavorable.

Prévoir la possibilité pour les collectivités territoriales de préempter des espaces en gare afin de développer certains services me paraît excessif. Cela pourrait conduire à désorganiser Cela pourrait conduire à désorganiser la gestion de ces espaces et à freiner le développement des recettes des gares résultant de l'installation d'activités commerciales. D'ailleurs, rien n'est précisé dans cet amendement sur les modalités d'une telle mise à disposition ni- et c'est le plus important - sur le loyer qui serait versé pour l'utilisation de tels espaces.

En commission, nous avons déjà prévu que les collectivités seront associées à la gestion des grandes gares ou ensembles de gares au travers de comités de concertation.

n° 36 tend à ce que le projet de contrat conclu entre l'État et Gares & Connexions sur des objectifs spécifiques à la gestion des gares soit soumis pour avis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental. Étant donné que le contrat pluriannuel qui sera conclu entre le gestionnaire de gares et l'État portera sur des objectifs relatifs à la trajectoire financière de Gares & Connexions ou aux prestations effectuées, il est indispensable qu'il soit soumis à l'ARAFER. En revanche, l'opportunité de soumettre ce projet pour avis au CESE et au Parlement est moins évidente. Bien sûr, cela va de soi, le Parlement a son mot à dire sur les grandes perspectives de développement des gares. Toutefois, il n'y a pas besoin de formaliser cette expression en avis pour que le Parlement se saisisse du sujet.

tend à ce que les accords collectifs qui seront négociés par les instances communes du groupe public unifié s'appliquent à l'ensemble des sociétés du groupe. À mon sens, il convient au contraire de faire confiance aux partenaires sociaux pour pour déterminer par voie d'accords collectifs les conditions du dialogue social au sein du groupe public unifié, ainsi que le niveau pertinent pour organiser la négociation sociale en fonction des thèmes abordés. Certains sujets auront vocation à être négociés à l'échelon de l'ensemble du groupe public, quand d'autres pourront faire l'objet d'une négociation décentralisée auprès de chaque entité. Il reviendra aux partenaires sociaux d'en décider. Je sollicite le retrait de cet amendement,

permettant de conforter la négociation sociale qui s'engagera dans les semaines à venir entre les organisations syndicales et la direction du groupe SNCF. L'unité sociale du groupe public unifié suppose en effet que les salariés de ces entités bénéficient d'un socle de

de prendre par voie réglementaire des mesures relatives aux conditions d'exercice du dialogue social au sein du groupe public unifié si les partenaires sociaux n'arrivent pas à adopter un accord collectif qui est prévu dans un délai de six mois. il faut quand même bien prévoir une solution en cas d'échec des négociations et d'impossibilité d'aboutir à un tel accord collectif. Cependant, sur ce sujet, comme sur d'autres, j'ai confiance en la capacité

inscrire l'inaliénabilité du capital dans le statut n'est pas plus protecteur que ce qui est prévu. L'avis est défavorable. Les de l'amendement n° 78 veulent inscrire dans les statuts initiaux des sociétés du groupe public unifié un mécanisme d'agrément pour la cession des actions détenues par l'État. Étant donné que l'article 1 A prévoit l'incessibilité des capitaux des entités du groupe, cet amendement me semble dénué de tout fondement. L'avis est défavorable. L'objectif poursuivi par les auteurs de l'amendement n° 76 est de maintenir les dispositions régissant le statut aux salariés employés après le 1 janvier 2020. En fait, il s'agit de s'opposer à la fin du recrutement au statut

vise à empêcher l'exercice des activités ferroviaires par le biais de filiales, ce qui reviendrait à empêcher Keolis, par exemple, d'avoir une activité ferroviaire, ce qu'elle a d'ores et déjà, en Allemagne notamment. L'avis est défavorable.

C'est une préoccupation que je partage et qui a conduit le Gouvernement à présenter devant la commission des amendements pour conforter l'unité sociale au sein d'un périmètre ferroviaire social unifié,

amendement. L'amendement n° 23 a pour objet de faire du recrutement au statut la norme et du recrutement à la convention collective l'exception. Comme vous le savez, le Gouvernement souhaite mettre fin au recrutement au statut au 1 janvier 2020, donc je suis défavorable

faire obstacle à la filialisation des gares. J'ai indiqué qu'il était important de donner une autonomie de gestion

souhaitent prévoir l'entrée de l'État, de collectivités locales ou d'autres acteurs publics dans le capital de Gares & Connexions. Cette hypothèse n'est pas envisagée par le Gouvernement, ce qui me pousse à donner un avis défavorable. n° 237, il s'agit de préciser la composition des instances de gouvernance de Gares & Connexions.

n° 129, le gestionnaire des gares serait sous le contrôle de son actionnaire exclusif et les comptes de la filiale seraient normalement consolidés par intégration globale dans les comptes de SNCF Réseau selon les principes comptables généraux. La loi n'a pas à prévoir de dérogation, mais je veux en revanche vous rassurer sur ce que je pense être votre préoccupation, préserver la capacité d'investissement de la filiale chargée des gares. Tout d'abord, l'autonomie de la filiale a été explicitée dans un amendement voté en commission. Il ne s'agira pas d'une simple direction de SNCF Réseau. Ensuite, la loi prévoit la définition d'un contrat pluriannuel conclu directement avec l'État. Enfin, la filiale n'entrera pas dans le champ de la règle d'or, qui vise à éviter un endettement excessif de SNCF Réseau. Avec ces différentes dispositions, vous avez toutes les garanties sur le fait que Gares & Connexions ne sera pas freinée dans ses besoins d'investissement, le cas échéant avec un endettement soutenable. Cette dérogation au code de commerce ne me semble pas nécessaire ni même souhaitable. L'avis est défavorable.

Il ne me semble pas de bonne pratique de demander un avis au Parlement, qui légifère et contrôle l'action du Gouvernement, mais qui n'est pas un organe consultatif susceptible d'exprimer un avis. Par ailleurs, une consultation du CESE n'entre pas dans son champ de compétences. Donc, l'avis est défavorable. n° 74 vise à empêcher toute possibilité de créer des filiales pour la SNCF.

pas. Le service public, depuis la décentralisation, est organisé par les régions, et non plus par la SNCF. Je pense que c'est une bonne garantie

les modalités du dialogue social à la nouvelle organisation du groupe SNCF. De la sorte, cet amendement les priverait de la faculté de définir le bon niveau de négociation en fonction des thèmes et en tenant compte des spécificités de chacun de ces niveaux. C'est pourtant une attente formulée par certaines organisations syndicales.

rectifié. Par cohérence avec leur amendement n° 149 rectifié , qui vise à supprimer la possibilité pour les partenaires sociaux d'adapter le cadre d'exercice du dialogue social,

de leur part -la possibilité de définir les conditions et le niveau de négociation les plus adaptés à la suite de la mise en place de la nouvelle organisation du groupe. Pour garantir le bon déroulement du dialogue social au sein de l'entreprise, il est nécessaire de prévoir un dispositif supplétif, de façon à inciter les partenaires sociaux à fixer les modalités de la négociation collective. Je suis donc aussi défavorable à cet amendement.

est de revenir sur l'arrêt du recrutement au statut au 1 janvier 2020. En réalité, vous êtes en train de perturber, si je puis dire, la clause de continuité sociale, qui est strictement celle qui avait été mise en place dans la LOTI,